Mon groupe se félicite de cette annonce, tant le fossé entre nos concitoyens et nos institutions judiciaires semble se creuser. Pourtant, la relation de confiance est essentielle pour légitimer les décisions qui sont rendues au nom du peuple français. Des jurisprudences récentes ont pu susciter l'incompréhension ou l'émotion dans l'opinion. Toutefois, dans un État de droit, la justice ne se confond pas avec la morale. Elle applique la loi :. Surtout, pour nous, républicains de tous bords, il n'y a pas à choisir comme d'aucuns l'ont fait entre forces de l'ordre et magistrats. Tous sont des fonctionnaires dévoués, qui font vivre le service public et défendent nos valeurs républicaines au quotidien. Je tiens à les saluer et à les remercier, et non à les opposer, au moment où nous devons renforcer notre cohésion nationale. Monsieur le Premier ministre, ce dont notre justice n'a pas besoin, c'est d'une énième consultation véhiculant son lot de promesses qui n'aboutiront pas, comme nous en avons trop connu, et qui décevront une nouvelle fois les professionnels du droit comme les citoyens. Pour notre part, nous défendons une justice plus accessible, plus simple et plus efficace. Monsieur le Premier ministre, comment entendez-vous restaurer la confiance entre nos concitoyens et notre justice ?

ne donne pas à la justice ses moyens d'intervention. Il en résulte que l'action des forces de l'ordre se trouve parfois sans suite et que des situations d'impunité peuvent être ressenties de manière inacceptable par certains de nos concitoyens, par les élus

le déploiement, dès 2021, de moyens nouveaux affectés au budget de ce ministère. Il s'agit, en particulier, de rendre plus rapide et effective la réponse judiciaire, d'améliorer la politique des peines, de garantir la dignité et la réinsertion des prisonniers et de moderniser le fonctionnement des juridictions. Mesdames, messieurs les sénateurs, c'est ce que nous nous attachons à faire.

Le Président de la République, précisément parce que le renforcement de l'autorité judiciaire et les moyens consacrés au service public de la justice sont au coeur de l'action de ce gouvernement, a décidé

que, dans une république démocratique comme la nôtre, la séparation des pouvoirs et le respect de l'État de droit doivent lier l'ensemble de nos concitoyens.

redonner à notre justice les moyens qui lui ont été trop longtemps comptés. La semaine dernière, nous avons eu plusieurs questions sur ce sujet, ici même, au Sénat,

selon lequel les États généraux de la justice ne doivent pas devenir « un lieu de pugilat politique ou électoraliste ». La parole est à M. Daniel Salmon, pour le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

nous apprenions que l'EPR de Taishan, en Chine, connaissait une augmentation de la concentration de certains gaz rares dans le circuit primaire de son réacteur n° 1. Les autorités chinoises se veulent rassurantes, le taux de radiation se situant dans les limites autorisées par les normes chinoises, limites toutefois trois fois supérieures aux normes françaises. Cette géométrie variable permet d'éviter l'arrêt du réacteur ... Mme la ministre Pompili tenait, mardi matin, les propos suivants à la radio : « Il ne faut pas qu'on ait une réflexion sur notre politique énergétique en partant d'un fait. » Certes, mais les faits sont têtus, ou plutôt les défauts et incidents s'accumulent depuis de nombreuses années ! À Flamanville, ont été pointées des défaillances sur le béton, les soudures, le pont polaire, les valves construites à l'envers, les piquages, ou encore les accidents du travail. Et je ne déroule pas toute la liste. À cela s'ajoutent les dérives financières : plus de 20 milliards d'euros en 2020, soit six fois plus que le coût initialement prévu, et un retard de livraison qui approche les dix ans. En Finlande, matériels et matériaux souffrent de défauts. Le retard de livraison est tel- plus de treize ans -que les équipements sont déjà trop vieux et doivent être remplacés. est de 7 milliards d'euros, dont près de 800 millions d'euros à la charge de l'État. En Angleterre, Hinkley Point connaît également retards et dérive des coûts. La Cour des comptes évoque, au sujet des EPR, un échec opérationnel, des dérives des coûts et des délais considérables. monde le sait, le coût du mégawattheure nucléaire est largement sous-estimé. À l'aune de ce que l'on peut qualifier de fiasco industriel, vous semble-t-il pertinent de poursuivre cet engagement à construire de nouveaux EPR,

et qu'ils sont exploités par une société chinoise, dont EDF est un actionnaire minoritaire et Framatome un prestataire. L'exploitation et la sûreté relèvent donc des autorités chinoises et de leur responsabilité souveraine. Il ne m'appartient pas de m'y substituer, même si, bien sûr, nos contacts sont fréquents. fréquents. Au-delà de la situation chinoise, vous posez la question du mix énergétique en France. La réponse est simple : notre politique énergétique est un mix avec diversification et résilience. Il n'est pas responsable de proposer aux Français une seule énergie, quelle qu'elle soit, comme solution au problème de la transition écologique dans notre pays. Tous les pays du monde font en sorte de ne pas dépendre d'une seule source d'énergie pour la production d'électricité. Nous avons besoin de solutions de rechange. Le nucléaire, comme toutes les énergies, présente des avantages : il est décarboné. Il présente également des inconvénients, parmi la gestion des déchets à long terme, mais aussi, peut-être de façon peut-être moins connue, la mobilisation des cours d'eau pour les opérations de refroidissement. C'est pour cela que nous avons l'intention de diminuer, d'ici à 2035, la part du nucléaire dans notre mix électrique, de 70 % à 50 %. À ce jour, le seul projet d'EPR que nous développons en France est celui de Flamanville. À la suite du rapport de la Cour des comptes, l'État a demandé à EDF de mettre en oeuvre l'intégralité des recommandations de l'audit conduit par Jean-Martin Folz. Folz. La diversification de notre mix reposera sur les énergies renouvelables : nous passerons à 25 % en 2020 et à 40 % en 2030, en développant, comme le prévoit la programmation pluriannuelle de l'énergie, le solaire, la méthanisation, l'hydrogène, l'éolien terrestre et maritime. Ces moyens nous permettront de produire une électricité qui restera, comme elle l'est aujourd'hui, l'une des plus décarbonées d'Europe. La parole est

Avec le soutien de ses partenaires, la France se bat pour faire reculer le terrorisme au Sahel. Néanmoins, la situation de la région se dégrade. Nous constatons que le nombre de victimes d'attaques terroristes reste élevé au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Des pays sont en train de s'enfoncer dans l'instabilité politique, et les djihadistes poursuivent leurs méfaits. La présence française est capitale pour la sécurité du Sahel. Le week-end dernier, un raid a permis de neutraliser et de capturer des cadres de l'État islamique. Notre armée continue de faire un travail remarquable. En 2023, après une sortie progressive, vous annoncez une présence réduite, avec deux objectifs : la formation des armées locales et la conduite d'opérations antiterroristes. Les parlementaires que nous sommes, qui ont toujours soutenu l'action française au Sahel, auraient souhaité être consultés sur le changement majeur de stratégie que constitue cette décision. Le retrait d'une partie de nos forces s'inscrit-il dans un programme stratégique concerté avec nos partenaires africains, européens et américains ? Sur quelles forces pourrons-nous compter pour lutter contre le terrorisme dans une région cinq fois plus étendue que l'Afghanistan ?

Je voudrais être très claire, tout d'abord en rappelant que nous sommes présents au Sahel à la demande des États du G5 Sahel. Par ailleurs, nous ne quitterons pas la région aux côtés de nos partenaires sahéliens, mais aussi européens et internationaux, notre engagement contre le terrorisme, qui reste notre priorité absolue. Ce que nous voulons, c'est changer de logique. Nous voulons aller vers davantage de coopération avec les Sahéliens et leur transférer progressivement la responsabilité des opérations. Avec nos partenaires européens, nous voulons aussi coopérer de façon encore plus étroite, pour les soutenir, par des formations et par de l'accompagnement opérationnel. nous souhaitons travailler avec les pays du golfe de Guinée, qui sont exposés, eux aussi, au risque d'extension de la menace terroriste. Cette évolution nous conduira à réorganiser notre dispositif de façon significative sur le plan militaire, en nous appuyant notamment sur la force Takuba, qui rassemble des détachements de forces spéciales européennes, en soutien aux forces locales. Les modalités et le calendrier de cette transformation de notre engagement seront précisés ultérieurement. Je réponds directement à votre question, monsieur le sénateur : nous allons d'abord consulter nos partenaires, puisque ce sont eux qui sont sur le terrain avec nous. Je voudrais souligner devant vous que tous nos interlocuteurs nous ont confirmé leur souhait de poursuivre la lutte contre le terrorisme. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir, mais cette coopération avec nos partenaires est la clé du renforcement de notre engagement collectif au Sahel contre le terrorisme. La

à lutter contre le djihadisme et le terrorisme islamiste partout dans le monde. Depuis des années, les gouvernements successifs ont dit à la Haute Assemblée que lutter partout dans le monde, c'était garantir l'intégrité du territoire français et la sécurité des Français en général. quelle est votre détermination à lutter, partout dans le monde, contre le djihadisme

internationale, singulièrement renforcé nos capacités et nos moyens de collaboration. Cette action signifie aussi l'intervention armée, quand c'est nécessaire. Nous le faisons au Sahel, et Mme la ministre des armées vient de confirmer cette orientation contre-terroriste de l'inflexion de notre organisation au Sahel. Nous le faisons aussi toujours en Syrie, par l'intervention de nos forces basées en Jordanie. Nous le faisons également les Nations unies, puisque, en ce moment même, est en train d'être définie la stratégie antiterroriste qui devrait réunir l'ensemble des États membres des Nations unies, sur la base d'éléments

d'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité, qui fixe des normes et prévoit des sanctions à l'égard de toute complicité sur le financement du terrorisme. Nous le faisons aussi en luttant contre la diffusion du terrorisme en ligne,

globale, régulièrement révisée au niveau national, dans les conseils de défense que tient le Président de la République.

etc. Par ailleurs, la Turquie n'hésite pas à dire qu'elle utilise des mercenaires djihadistes syriens contre l'Arménie, contre les Kurdes, en Afghanistan ou en Libye. Nos amis arméniens, nos amis kurdes, nos amis libyens, auprès de qui nous intervenons pour que la démocratie soit rétablie, se demandent où est l'Europe et où est la France. Bien sûr, nous protestons ! Bien sûr, nous nous indignons ! Mais c'est insuffisant pour préserver la liberté de ces peuples menacés. Lorsque l'Europe et la France ne défendent pas avec suffisamment de fermeté les valeurs démocratiques, lorsque notre jeu diplomatique, notamment par rapport à la Turquie, n'est pas d'une netteté absolue- c'est le moins que l'on puisse dire ces derniers jours -, nous remettons en cause nos propres valeurs de liberté et de démocratie. J'espère que nous n'en paierons pas un jour le prix.

élections législatives partielles, la distribution de la propagande électorale a été catastrophique dans les territoires où elle devait être effectuée par la société Adrexo, qui a remporté l'appel d'offres de l'État pour 51 départements. Les 20 et 27 juin prochain ont lieu les élections départementales et régionales, et l'on note déjà des dysfonctionnements : des envois prématurés ou qui n'arrivent pas, et, pis encore, des défauts de distribution, avec des enveloppes jetées par paquets, soit dans une même boîte aux lettres, soit dans des poubelles. Alors que l'abstention atteint des niveaux record, nous prenons le risque de voir certains électeurs privés d'informations essentielles. Pourquoi avoir retiré une partie du marché à La Poste, qui assure pourtant le service public de distribution du courrier toute l'année dans notre pays ? Elle seule possède l'adresse cartographiée de tous les Français, parcourt chaque jour notre territoire et connaît chaque boîte aux lettres. Par ailleurs, le traitement différencié des élections départementales et régionales est inacceptable et donne l'impression qu'il y aurait une petite et une grande élection. Pourquoi différencier les délais de remise des professions de foi entre les élections départementales et les élections régionales, qui auront pourtant lieu à la même date ? Cette désorganisation perturbe les électeurs, avec une propagande reçue soit trop tôt, soit trop tard, ou non reçue. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous garantir que l'ensemble des électeurs auront les informations nécessaires pour aller voter les 20 et 27 juin prochain ?

au moment des premier et second tours. Le code électoral, contrairement à ce que je peux entendre, n'a jamais prévu un temps de distribution. Oui, il y a eu des envois faits trois semaines avant le premier tour.

cette demande est défendue par des militants syndicaux, associatifs et politiques, notamment dans les pays pauvres, qui se mobilisent contre les effets de la propriété intellectuelle sur le droit à la santé et l'accès effectif aux soins et aux produits pharmaceutiques. Après avoir refusé la levée des brevets, le Président de la République a indiqué, mercredi dernier devant des représentants d'associations, et, jeudi, en conférence de presse, que la France soutiendrait la demande de l'Afrique du Sud et de l'Inde. Néanmoins, des ambiguïtés demeurent. Monsieur le ministre, alors qu'une réunion informelle doit justement se tenir demain à l'OMC, pouvez-vous nous préciser la position de la France sur ce sujet ? Quelles sont les modifications que le Président de la République souhaite apporter, à la demande de l'Afrique du Sud et de l'Inde ? La parole nous sommes tout à fait convaincus de la nécessité de faire du vaccin un bien public mondial. Cet objectif requiert un certain nombre de conditions : des contributions financières

pour élaborer la mise en oeuvre du projet d'usine de vaccins en Afrique, singulièrement en Afrique du Sud et au Sénégal. L'objectif est de faire en sorte que soient levés le plus

J'ai bien noté que, jusqu'à présent, les États-Unis d'Amérique, tout en étant favorables à la levée des brevets, ne l'étaient pas à celle des processus d'exportation. Il semble que cette donnée soit en train de changer depuis la réunion du week-end dernier, et c'est tant mieux. En ce qui concerne les brevets,

l'accaparement des brevets par les entreprises de production pharmaceutique. Il s'agit simplement de les mettre en oeuvre. L'Union européenne vient de formuler une proposition en ce sens.

Sud et l'Inde attendent des actes, non des paroles Madame la secrétaire d'État, en 2019, mon département de l'Eure avait été l'un des treize départements pilotes pour la première édition du service national universel, le SNU. Le SNU est encore aujourd'hui en phase d'expérimentation, et un bilan d'étape paraît nécessaire avant d'envisager sa généralisation. Vous êtes sur le point de lancer les séjours de cohésion, pour la première fois dans tous les départements du pays, du 21 juin au 2 juillet prochain. L'un des intérêts incontestables du SNU est qu'il constitue un rite de passage vers la citoyenneté, à l'heure où les valeurs de notre République sont parfois très mises à mal. Par ailleurs, il permet aux jeunes de découvrir un autre territoire et favorise le brassage de jeunes d'horizons et de milieux sociaux très différents. À ce titre, lorsqu'elle fut auditionnée par le Sénat le 4 mai dernier, Emmanuelle Pérès, la déléguée interministérielle à la jeunesse, a déclaré qu'il fallait encore renforcer cette mixité sociale- c'est essentiel. Enfin, un tel dispositif paraît d'autant plus opportun aujourd'hui que la crise sanitaire a fragilisé le marché du travail et l'employabilité des jeunes : le SNU apparaît comme un outil pour créer un pont vers l'emploi.

les soignantes et les soignants étaient hier dans la rue pour réclamer des revalorisations salariales et l'augmentation de leurs effectifs. Le collectif « Notre hôpital, c'est vous » a dévoilé ses propositions pour remettre l'hôpital public réellement au service au service de la santé des Françaises et des Français. Voilà ce qu'il rappelle : l'égal accès aux soins doit être assuré par le service public ; il faut augmenter le nombre de soignantes et soignants

les citoyennes et les citoyens définissent la stratégie sanitaire et délibèrent sur ses moyens humains et financiers. La santé est la préoccupation majeure dans notre pays. Les propositions du collectif sont pleinement à la hauteur de cet enjeu. Elles tournent la page des fermetures de maternités et des longs trajets en ambulance pour consulter des spécialistes. Elles font oublier l'extrême fragilité du système hospitalier, qui a dû répondre tant bien que mal à la crise sanitaire depuis quinze mois. Nous, apportons tout notre soutien à cet appel et appuyons la démarche du référendum d'initiative partagée. Je salue l'engagement de notre collègue Bernard Jomier aux côtés de ce collectif. Ma question est simple : qu'attendez-vous pour engager cette refonte du système de santé, qui placerait,

Le Sénat sait bien que le fameux Ségur- je pourrais parler du volet investissements, mais vous m'interrogez à bon droit sur le volet humain -résulte d'une négociation et d'un accord majoritaire conclu avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur. J'y insiste parce que, au-delà du fond, cette méthode me semble extrêmement importante. La parole

Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur. Très récemment, le Président de la République a annoncé qu'il entendait renforcer les mesures de lutte contre l'immigration clandestine, notamment en augmentant le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire national. Le dernier avis budgétaire de la commission des lois

Vendredi dernier, le rapporteur public du Conseil d'État a estimé insuffisantes les mesures pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il rejoint en cela l'avis de bon nombre d'instances comme le Conseil national de la transition écologique, le CNTE, et le Haut Conseil pour le climat, qui vous rappellent que la décennie en cours est cruciale

Êtes-vous prête à enrichir votre texte au Sénat de dispositions rehaussant nos ambitions ? Le travail que nous allons effectuer pendant les dix prochains jours est-il condamné à disparaître en commission mixte paritaire ? Madame la ministre, ma question est simple : après avoir redéfini à la baisse notre trajectoire bas-carbone, et considérant, comme vous l'avez reconnu à plusieurs reprises, que ce projet de loi ne suffira pas, quand allez-vous proposer au pays un véritable plan de décarbonation de l'économie et un calendrier de réformes conforme à nos engagements nationaux et européens ?

Si je vous interpelle aujourd'hui, c'est parce que le compte n'y est pas, comme l'a souligné la Convention citoyenne pour le climat. Je comprends donc, madame la ministre, qu'il est important pour vous d'attendre un énième Grenelle ou un nouveau Varenne avant d'être tancée d'agir par le Conseil d'État. Vous mettez la France en état d'insécurité environnementale, alors que le quinquennat précédent nous avait placés à la pointe du écologique. Vous pouvez encore relever l'ambition de ce texte en matière de rénovation énergétique des logements, de transports, de transition agroécologique en suivant nos propositions. Faites en sorte que le projet de loi Climat ne soit pas qu'une goutte d'eau comparée à l'océan des besoins. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, « gouverner, c'est prévoir ». Cet adage, que le Gouvernement devrait réciter sans cesse, s'applique à toutes les politiques publiques, notamment dans le domaine médico-social. âgées dépendantes, est extrêmement préoccupante. Déjà, avant la crise du covid, le personnel, souvent en sous-effectif, était en souffrance, et beaucoup d'établissements devaient investir dans le cadre de travaux d'humanisation et de rénovation. La crise sanitaire que nous avons connue a très largement amplifié cette situation. De nombreuses réorganisations sont nécessaires dans les structures. De plus, à la suite de la pandémie, les préconisations formulées par les ARS, les agences régionales de santé, imposent sas de décontamination, accès dédiés, unités autonomes ... -qui représentent des coûts élevés et nécessitent des surfaces de construction plus importantes. Parallèlement, dans ce contexte, l'application du décret éco-énergie tertiaire au secteur médico-social imposera de nouvelles normes environnementales, donc de nouveaux coûts d'investissement. Nous ne remettons pas en cause la pertinence des mesures liées au covid, ni celle des actions en faveur de la rénovation énergétique, mais l'impact financier et le calendrier imposé semblent intenables Des enveloppes budgétaires sont prévues dans les mesures du Ségur immobilier, mais seront-elles suffisantes au regard des enjeux imposés ? Ma question est simple : avez-vous évalué- pour prévoir -les besoins sur l'ensemble du territoire national ? Quels sont-ils ? Quels moyens et quelles aides seront proposés par l'État ?

Monsieur le ministre, lors d'une crise sanitaire, il est crucial que des enquêtes scientifiques complètes et transparentes puissent être menées. Nos concitoyens ont le droit de connaître l'origine d'une pandémie qui a durement affecté leur vie quotidienne- c'est un doux euphémisme. En janvier En janvier dernier, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a mené l'enquête en Chine pour comprendre comment le virus de la covid-19 avait été transmis à l'homme. Toutefois, il semblerait que cette organisation n'ait pu travailler librement lors de ce séjour de quatre semaines à Wuhan. Les résultats des experts sur place étaient, semble-t-il, surveillés de près, même de très près ; leurs conclusions devaient être approuvées par un groupe de travail, sous l'autorité directe du gouvernement chinois On le voit, on le sent, on le sait, l'information est contrôlée, filtrée et probablement censurée. Plusieurs journalistes chinois ont d'ailleurs été arrêtés lorsqu'ils ont eu l'outrecuidance de sonner l'alarme à propos du virus. Or les citoyens chinois et ceux du monde entier ont droit à la vérité sur l'origine de cette pandémie. Ce problème de transparence est d'ailleurs d'actualité : à la suite d'un incident technique survenu avant-hier sur l'un des réacteurs nucléaires de la centrale de Taishan, dans le sud-ouest de la Chine, l'exploitant de la centrale s'est contenté laconiquement de déclarer que les indicateurs environnementaux étaient « normaux », sans autre précision. Le ministère chinois des affaires étrangères n'est guère plus loquace sur le sujet.

... -, une mission de l'OMS s'est rendue en Chine, pour essayer d'identifier l'origine de la covid-19 et de comprendre les mécanismes de transmission du virus. Le rapport de cette première mission a été remis voilà quelques mois. C'est une étape importante

étape. Nous considérons que le travail scientifique doit se poursuivre dans la plus grande transparence et nous appelons l'ensemble des États membres, à commencer par la Chine, à la collaboration la plus étroite

Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous venez d'annoncer la levée anticipée du couvre-feu ; c'est là une décision bienvenue au regard de la situation sanitaire et des huit mois de limitation de nos libertés qui viennent

respectaient scrupuleusement le couvre-feu et quittaient la terrasse du Dock 713, guinguette en bord de Loire, à vingt-trois heures, au même moment les privilégiés des loges de Roland-Garros scandaient « Merci Macron, merci Macron ! » en hommage à celui qui les avait autorisés à ne pas respecter le couvre-feu. Quelques instants plus tard, aux Invalides, des jeunes se faisaient charger pour non-respect dudit couvre-feu ... Ce « en même temps » a été vécu comme une injustice devant le fait du prince : « Selon que vous serez puissant ou misérable ... » Ce week-end, nos concitoyens ont vu en boucle les images de vos ministres. Ils ont vu votre ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur chanter en meeting sur une estrade, sans masque ! Ils ont vu le ministre de l'intérieur,

Monsieur le Premier ministre, à quatre jours des élections départementales et régionales, après le baiser qui tue dans le Sud et le parachutage des ministres dans le Nord, nos concitoyens s'interrogent votre gouvernement cherche-t-il ce faisant, de façon volontaire, mais irresponsable, à susciter l'incompréhension et la colère des Français, pour mieux la faire exploser dans les urnes ? La parole est à M. le ministre de l'intérieur. Devant une

je me dis que c'est la politique des grincheux qui vous satisfait. Ne pouvez-vous pas vous réjouir que les Français soient manifestement heureux de revivre et que, oui, les mesures mises en oeuvre par le Gouvernement soient de bonnes mesures ? Vous avez parlé de Roland-Garros.

dans le même temps, ce geste a été ressenti comme une gifle par toutes celles et tous ceux que l'on a appelés les « oubliés du Ségur » : tous les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes, qui exercent pourtant les mêmes métiers, avec les mêmes diplômes et sous le même statut, ont été tenus à l'écart de ce processus. L'une des premières conséquences a été une perte d'attractivité de certains de ces métiers. Mon collègue Franck Montaugé me disait hier soir encore avoir été interpellé par des soignants du secteur privé de l'accompagnement spécialisé, qui lui disaient quitter leurs structures « la boule au ventre », pour aller chercher quelques dizaines d'euros supplémentaires dans le secteur qui a bénéficié du Ségur. Après avoir bataillé de longs mois, certains de ces oubliés ont enfin été entendus. À partir du 1 octobre prochain, ils bénéficieront de ce même complément. En avril dernier, ma collègue Michelle Meunier vous interpellait déjà sur les « nouveaux oubliés » que le Gouvernement était en train de créer en répondant au compte-gouttes aux légitimes demandes des différentes professions de la chaîne du soin. Le plus inquiétant est que vous persistez dans cette politique de division, qui a causé tant de sentiments d'injustice et de désorganisation dans ce secteur. Ainsi, la revalorisation consentie le 28 mai ne se fera en définitive que pour les établissements bénéficiant d'un financement de l'assurance maladie- c'est grave ! Sont donc laissés de côté tous les personnels des établissements relevant du financement des conseils départementaux. C'est pourtant la solidarité nationale qui doit jouer, d'autant que les inégalités entre départements peuvent être grandes. Le département dont je suis l'élu, celui de la Loire, est l'un des deux seuls de France à avoir refusé de verser la prime covid aux personnels des services de soins et d'aide à domicile.

Dans le cadre des accords du Ségur, vous l'avez dit, une augmentation de 180 euros net par mois avait été décidée pour 1,5 million de professionnels des établissements de santé et des Ehpad. Cette augmentation est inédite et méritée ; elle concerne également plus de 90 000 professionnels qui exercent leurs fonctions auprès de personnes en situation de handicap de personnes âgées ou en difficulté sociale. Récemment a été signé un accord de méthode relatif à l'attribution d'un complément de rémunération aux personnels soignants des structures pour personnes handicapées et des services de soins à domicile. Cet accord a été conclu

examinée à la rentrée prochaine par votre assemblée. Les organismes gestionnaires privés non lucratifs pourront, s'ils le souhaitent, en anticiper le versement. Cet accord a également permis de tracer des perspectives cruciales. Il s'agit désormais d'établir, selon un calendrier de la revalorisation des autres métiers de l'accompagnement et du médico-social, dont les situations ne sont pas identiques, mais qui tous jouent un rôle indispensable dans l'accompagnement des plus fragiles. Les parties prenantes devront faire émerger des propositions adaptées pour ces secteurs, au regard de la réalité de de leurs conditions globales de rémunération, notamment. L'État apportera une contribution financière en fonction des propositions qui seront faites. Il importe, dans tous les cas, que l'ensemble des leviers soient activés pour garantir l'attractivité des métiers du soin et de l'accompagnement. Un premier point sera fait avec l'ensemble des signataires de l'accord avant l'été, mais c'est surtout d'ici

a répondu présent en votant les lois de finances rectificatives successives pour 2020. Toutefois, en 2021, alors que la croissance est de retour selon vos prévisions,

Une dette de la sécurité sociale qui, pour la première fois dans l'histoire, sera supérieure à la dette d'investissement des collectivités locales ! Le ministre de l'économie nous dit qu'il faudra bien en finir avec le « quoi qu'il en coûte ». Le ministre du budget abonde en son sens. Ils se font taper sur le bec, parce qu'il faut continuer

n'aurait-on entendu aujourd'hui si nous n'avions pas accompagné les entreprises ?

qui les attendent, au moment où s'ouvre la phase complémentaire d'admission sur la plateforme Parcoursup pour les quelque 168 000 candidats qui n'ont toujours pas de proposition d'affectation.

assez largement, et même au-delà du raisonnable, puisque certains professeurs confient avoir très grandement surnoté dans le cadre du contrôle continu, qui pèse si lourdement cette année. Résultat : de très bons élèves, dont le dossier est excellent, se retrouvent sans aucune proposition d'affectation, une forme de suspicion quant à la transparence du processus de sélection et d'admission. Ces bons élèves, à qui la République promettait de récompenser le mérite et le travail, sont totalement désemparés face à cette situation qu'ils estiment évidemment injuste.

permettez-moi de tirer profit de votre question pour revenir sur l'avancée de cette procédure et, avant toute chose, pour souhaiter bonne chance à tous les jeunes qui vont passer le baccalauréat cette année. Vous mentionnez le cas de très bons profils qui n'auraient pas obtenu les propositions de leur choix. Il me semble important de le répéter, depuis le 27 mai tous les candidats qui n'ont fait de demandes

demande qu'une attention toute particulière soit apportée « à la manière dont ces formations veillent à conserver dans leurs classements une diversité de profils, ainsi qu'aux efforts qu'elles feront en matière d'ouverture sociale et d'équilibre de genre ». Cela ne peut que nous interroger, madame la ministre. Si ces critères sont intégrés aux algorithmes locaux, il serait bon que les candidats, leurs familles et, pourquoi pas, la représentation nationale en soient informés. Nous

La séance est reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents, réunie ce jour, sont consultables sur le site du Sénat.

été amoindri, il faut aussi le dire, par l'Assemblée nationale, voire- le terme est peut-être un peu fort -carrément dévoyé par le décret d'application, qui l'a ouvert, bien au-delà des associations et des entreprises de l'ESS, à toutes les entreprises du secteur, alors que l'objectif était justement de soutenir l'économie sociale et solidaire.

Il est donc apparu qu'il était indispensable de préciser la loi pour obtenir la modification du décret. Tel est l'objet de cet article 13 , et de cet amendement, qu'il fallait encore ajuster,

La version adoptée par la commission ne permet de répondre que partiellement au problème de rédaction que posaient le texte de la loi AGEC et son décret d'application, dans la mesure où elle conserve l'obligation

ouverts à l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire et ne fassent pas l'objet de procédures sélectives de type appel à projets. La loi anti-gaspillage avait en effet prévu que ces fonds pour le réemploi tiennent compte de deux critères seulement : le principe de proximité, d'une part, et, d'autre part, le critère ESUS, correspondant aux entreprises solidaires d'utilité sociale du code du travail. du travail. Or les études préparatoires menées en amont du déploiement de ces fonds, notamment pour les filières des équipements électriques et électroniques, des jouets et des articles de sport, ont montré que les critères retenus dans la loi anti-gaspillage, trop restrictifs, n'englobaient pas l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire

par les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors que 70 % des déchets produits chaque année en France sont issus du secteur de la construction et de la déconstruction,

Cette filière remet sur le marché des matériaux de construction à prix solidaire, permettant aux ménages précaires d'avoir accès à des matériaux de qualité pour des travaux de construction ou de rénovation. Ces structures ont en outre un rôle social dans les territoires, la mise en place de parcours d'insertion de personnes éloignées de l'emploi. Il apparaît donc essentiel de les soutenir et de et de réserver les financements de la filière à responsabilité élargie des producteurs relative aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment aux associations et entreprises de l'économie sociale et solidaire.

réunis au sein d'ESS France. Il vise à clarifier les choses en précisant que les financements sont attribués par ces fonds sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande, et sans avoir recours à des procédures sélectives de type appel à projets. Il tend par ailleurs à réserver les financements aux associations et entreprises de l'ESS.

il est apparu, lors de l'écriture du décret, que la rédaction adoptée à l'époque de la loi anti-gaspillage était un peu trop restrictive et ne permettait pas de répondre à l'intention initiale du législateur.

c'est important -en tant qu'anciennes parlementaires attachées au respect de la volonté du législateur, à faire évoluer la loi AGEC pour que l'ensemble de l'économie sociale et solidaire puisse véritablement bénéficier de ces fonds pour le réemploi. C'est donc un avis très favorable

Le développement du commerce en ligne, qui s'est beaucoup accru ces derniers temps à cause de la pandémie, a des effets pour le moins importants. La massification des importations de certains produits- électroniques, textile-habillement, jouets -dégrade l'empreinte carbone de la France. Nous connaissons une explosion des livraisons express et des livraisons à domicile, avec comme conséquence la multiplication des petits trajets entre les points de dépôts et les domiciles des particuliers- c'est ce que l'on appelle le dernier kilomètre -, qui intensifient les flux et détériorent la qualité de l'air- des émissions de gaz à effet de serre et de particules fines -, notamment au coeur des grandes villes. Cela entraîne aussi la croissance de la consommation d'emballages, ce qui dégrade encore le bilan carbone du commerce en ligne. Le développement du e-commerce a donc un coût environnemental de plus en plus important, ce qui nécessite des mesures pour réduire ses impacts nocifs sur la santé et l'environnement. s'ajoute le fait que le commerce en ligne engendre davantage de retours par rapport aux canaux traditionnels de la distribution, tout particulièrement dans le domaine du textile. Comme le souligne le rapport de l'inspection générale des finances, publié en février des finances, publié en février 2021, « le commerce en ligne présente un taux de retour important, estimé à environ 10 % sur la base des éléments communiqués à la mission et qui peut atteindre jusqu'à 30 % dans certaines filières comme le textile ». Ces retours impliquent de nouveaux trajets entre les entrepôts, les lieux de production et les services après-vente, pour les produits défectueux. Or la plupart de ces marchandises retournées à leur distributeur seraient non pas remises en vente, mais de nouveau exportées vers d'autres pays, pour y être détruites. Ainsi, Amazon aurait détruit 3,2 millions d'objets neufs selon une enquête du magazine. De telles pratiques seraient courantes dans le secteur du textile et de la mode. Elles contribuent à accroître l'empreinte carbone de la France et détériorent le bilan carbone du commerce en ligne, raison pour raison pour laquelle elles doivent être prohibées. Cet amendement vise à interdire la destruction ou l'exportation pour destruction des marchandises neuves du secteur de l'habillement et du prêt-à-porter, que le client a retourné au distributeur ou à la plateforme de vente en ligne. Quel

Cependant, la loi AGEC prévoit en son article 35 que les producteurs ou distributeurs sont tenus de réutiliser ou de recycler leurs invendus non alimentaires- un périmètre qui comprend donc les retours de textiles. Ce même article prévoit un régime de sanction adapté. Sur le plan législatif, cet amendement est satisfait. La loi étant entrée en vigueur depuis peu, il me semble pertinent de pouvoir d'abord tirer un premier bilan avant d'envisager une évolution des dispositions à cet égard.

des pièces détachées visibles pour l'automobile. Il permettra également de diminuer le coût de la réparation des automobiles et de favoriser la compétitivité des entreprises françaises, dans l'intérêt conjoint des consommateurs et des constructeurs. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis favorable.

effet de serre en 2030. Régulièrement dénoncée pour son opacité et son rôle dans les stratégies d'optimisation fiscale des grandes entreprises, la fiscalité avantageuse en faveur de la recherche est loin loin de concourir au développement de la recherche environnementale. Il apparaît donc nécessaire de mettre la stratégie nationale de soutien à la recherche française au service des mutations économiques et écologiques de demain.

Vous faites clairement principalement référence ici, monsieur le sénateur, au crédit d'impôt recherche, mesure générale qui contribue très directement à la compétitivité du territoire français pour les activités de recherche, mais aussi d'innovation. Il concerne, vous le savez, toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité et quelle que soit leur taille. J'ajoute que le cadre européen ne permet pas de discriminer en fonction des secteurs d'activité ou des thématiques de recherche. Le crédit d'impôt recherche ne découle pas de la stratégie nationale de recherche, la SNR ; il n'y a d'ailleurs aucun lien direct entre la SNR et le crédit d'impôt recherche. nationale fixe des orientations ; le crédit d'impôt est bien plus large : il sert toute la recherche et pas uniquement celle qui relève de la SNR, ce qui est plutôt une bonne chose pour notre tissu

un pays qui a confiance en son avenir investit dans la recherche. La recherche publique et privée est sans nul doute un levier déterminant dans la transition écologique, même si la réponse

process industriels moins consommateurs de matières premières et moins énergivores. L'article 14 de ce projet de loi manque d'ambition et se limite à une mise en cohérence de la stratégie nationale de recherche avec la stratégie bas-carbone, ainsi qu'avec la stratégie nationale pour la biodiversité et la programmation pluriannuelle de l'énergie.

l'octroi du crédit d'impôt recherche à des critères d'écoconditionnalité, mais d'utiliser le fait que la stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en oeuvre font l'objet d'un rapport biennal de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Opecst, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée,

Premièrement, il faut accorder la priorité aux dépenses publiques et aux incitations fiscales susceptibles de contribuer à soutenir la croissance potentielle, en particulier dans l'innovation, la recherche, l'industrie et le développement des compétences. Deuxièmement, toujours selon la Cour des comptes, il faut accélérer la transition écologique.

On ne peut pas nier l'engouement pour ce dispositif on ne peut plus avantageux, puisque les 26 360 entreprises bénéficiaires ont presque triplé depuis 2007, pour une absence de résultats. Un dernier avis de la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation, la Cnepi, publié en juin dernier, finit d'étayer la nécessité de supprimer le dispositif : pas d'impact significatif sur la probabilité de déposer un brevet, pas d'impact sur la valeur ajoutée des entreprises bénéficiaires, pas d'effet causal sur le taux d'investissement global des entreprises, pas d'effet significatif établi en ce qui concerne les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, et les grandes entreprises. Les impacts positifs ne se transforment de manière significative que sur certains indicateurs de performance économique- chiffre d'affaires, masse salariale et investissements incorporels -, mais rien de tel n'apparaît sur d'autres valeurs ajoutées- emploi ou exportation. Bref, nous souhaitons plus que jamais la suppression de cette niche fiscale, qui coûte beaucoup d'argent aux finances publiques. Le présent amendement est plus modeste. Il vise à reprendre une proposition de la Convention citoyenne pour le climat qui tend à interdire la perception de l'argent public au titre du CIR pour des activités liées à des énergies fossiles. Les dépenses de recherche visées par l'interdiction sont relatives tant à la prospection qu'à l'exploitation, au transport, à la distribution et à la consommation d'énergies fossiles. Comment concevoir, dans la situation de détresse climatique qui menace l'humanité dans toutes ses composantes,

l'amendement n° 788, la conditionnalité du crédit d'impôt recherche aux activités économiques contribuant à des objectifs environnementaux conduirait à une restriction importante du crédit d'impôt et pourrait conduire à un affaiblissement de la recherche française. L'avis de

de l'amendement précédent. Le CIR est une mesure générale, qui concerne toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille. Je rappelle aussi que le cadre européen ne permet pas de discriminer en fonction de secteurs ou de thématiques de recherche.

la nécessité d'une forte dimension d'investissement écologique : c'est écrit noir sur blanc dans la loi. J'ajouterai,

car notre pays a besoin d'accroître son effort de recherche. Nous ne sommes pas au niveau des objectifs que nous nous étions fixés ; je pense notamment à la stratégie de Lisbonne qui visait à ce que 3 % du PIB soit dédié à la recherche.

et d'inciter le maximum d'acteurs à investir dans ce domaine. C'est par des incitations, notamment fiscales, que l'on arrivera à mobiliser tout le monde et à faire en sorte que notre pays soit attractif pour tous ceux qui veulent entreprendre, rechercher et trouver. Je mets

La transition climatique ne pourra se faire sans les entreprises. Afin de piloter cette transition, celles-ci ont besoin de normes portant sur leur durabilité ; il s'agit d'échapper aux normes anglo-saxonnes. de prévoir sont en voie d'élaboration et d'harmonisation à l'échelon européen. Le projet de directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises a été présenté par la Commission européenne L'élaboration au sein de l'Union européenne des normes en matière de durabilité doit être articulée de manière cohérente avec la normalisation de l'information financière. Cette cohérence nécessite que les normalisateurs comptables nationaux, comme l'Autorité des normes comptables (ANC) en France, soient en mesure de contribuer à la réflexion européenne en cette matière.

pour confier à son comité consultatif, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par le décret n° 2010-56 du 15 janvier 2010, une compétence dans le domaine de l'information en matière de durabilité des entreprises. Quel est l'avis de la commission

l'ordonnance qui crée l'ANC, pour confier à son comité consultatif la mission de produire des avis et des prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des normes européennes et internationales relatives à la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises. La directive sur le de

élabore des normes techniques en la matière. Ces normes devront être étroitement articulées avec les normes comptables existantes relatives à l'information financière. Dans ce contexte,

Chacun sait également que les collectivités locales représentent, à elles seules, 70 % de l'investissement public. Inscrire 100 % de la commande publique dans les principes du développement durable, certes, c'est s'assurer de la durabilité des produits et de leur impact environnemental, mais c'est aussi renforcer la prise en compte de critères sociaux au service d'une société inclusive. Je pense tout particulièrement à une meilleure prise en compte dans les critères d'attribution de la part exécutée

Il est en effet réellement important de prendre en considération les aspects environnementaux dans la commande publique ; ce n'est pas un membre de la commission du développement durable qui dira le contraire ... Cependant, cela sera mis en place par des décrets d'application qui, eux, échapperont à l'analyse parlementaire. Or il est crucial de connaître les critères qui permettront de décider quelle entreprise est plus méritante qu'une autre d'un point de vue environnemental. La mise en pratique de cet article soulève de nombreuses incertitudes. Pour la commission d'appel d'offres, pour celui qui écrit le marché public ou celui qui va l'attribuer et le juger, il est relativement facile de démontrer, face à un critère de prix, quelle entreprise est la moins chère. En revanche, il est beaucoup plus difficile de juger et, surtout, de vérifier quelle entreprise a le plus faible impact environnemental. Les acheteurs publics attribuant les marchés- un montant de 200 milliards d'euros a été évoqué -ont besoin d'outils spécifiques, clairs, précis, pour être en mesure d'appliquer Quel sera le garde-fou pour que le bon sens de cet article ne se heurte pas aux barrières du droit de la concurrence et au nombre de contestations qui risquent de se faire jour ? J'espère que les discussions qui s'ouvrent sur cet article éclaireront ma lanterne.

Très tôt, elle a été identifiée comme un levier pour la reprise économique. Cela s'est traduit dans le plan de relance, qui prévoit un certain nombre de crédits pour inciter les collectivités à recourir massivement à l'investissement. Les enjeux autour de la commande publique sont en effet considérables.

depuis une dizaine d'années. Elle s'adapte progressivement aux défis contemporains : dématérialisation, souplesse, intégration de critères sociaux et environnementaux ... Depuis 2017, des mesures ont été adoptées pour faciliter l'accès à la commande publique. De nouvelles dispositions législatives et réglementaires

des nouveaux cahiers des clauses administratives générales et techniques (CCAG). Le texte que nous examinons poursuit, au travers de son article 15, cette volonté de faire des acheteurs publics des acteurs de la transition. Il est ainsi prévu d'imposer, dans les marchés publics et les concessions, les considérations liées aux aspects environnementaux des travaux, services ou fournitures achetés. Parallèlement à ces débats, ma collègue députée Sophie Beaudouin-Hubiere et moi-même avons mené près d'une cinquantaine d'auditions dans le cadre de la mission temporaire qui nous a été confiée par le Premier ministre. Celle-ci doit permettre de définir de nouvelles méthodes et outils afin d'inciter les collectivités à mieux prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans le cadre de leurs appels d'offres. Nous souhaitons développer la culture de l'évaluation au sein de la commande publique, en l'intégrant au baromètre de l'action publique et en développant des indicateurs clairs et lisibles par tous, ce qui permettra à chacun d'évaluer la politique d'achat de l'État et des collectivités locales.

ainsi que les membres de notre commission, qui ont largement contribué à améliorer le texte. Sur l'initiative de plusieurs groupes, nous avons assuré une meilleure prise en compte des objectifs du développement durable dans les achats publics. Nous avons également souhaité que les dispositions relatives au contrat de concession fassent l'objet d'une entrée en vigueur anticipée, à deux ans, considérant la spécificité de ces achats publics. Nous avons aussi contribué à renforcer la prise en compte des considérations relatives à l'insertion et à l'inclusion, dans le respect des limites posées par le droit européen de la commande publique. Nous avons beaucoup avancé, mais j'aurais souhaité aller plus loin sur ce sujet qui me tient tout particulièrement à coeur. Nous sommes cependant résolus à ne pas introduire de dispositions contraires au droit de l'Union européenne, dans un esprit de responsabilité pour nos collectivités territoriales. Je rappelle que, en matière de commande publique, l'insécurité juridique peut être lourde de conséquences. Des dispositions contraires au droit européen fragiliseraient l'ensemble des achats publics réalisés par nos collectivités territoriales.

raisonnable. L'examen à l'Assemblée nationale a ouvert la discussion de l'article 15 sur le sujet de la place du critère social. Au cours des débats, auxquels j'ai eu le plaisir de participer, j'ai eu l'occasion d'expliquer en détail pourquoi, en l'état des rédactions, nous ne pouvions y souscrire. Pascal Martin, avec l'appui de la commission des lois et de celle de l'aménagement du territoire et du développement durable, a souhaité revenir sur ces rédactions en prévoyant d'autres dispositions visant le même objectif.

nos entreprises, nos TPE et PME, mais aussi les acheteurs, les collectivités locales et, par construction, nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à la rédaction proposée par la commission, qui pose le principe d'un lien

appuyer cette transition écologique, mais aussi sociale, sur le territoire. Les députés ont souhaité renforcer l'obligation de publication de ces schémas. Le Gouvernement évolue dans ses réflexions. Ainsi, les consultations qu'il a menées permettent de penser qu'une publication annuelle sera utile pour accroître la dynamique et mobiliser un effet d'entraînement. Nous aurons sans doute l'occasion d'évoquer la meilleure prise en compte des ESUS dans les Spaser, et ce en parfaite cohérence avec l'objectif du Gouvernement de favoriser l'insertion par la commande publique. Il y a la loi et il y a son application. Pour accompagner cette application et accroître cette ambition, le Gouvernement est pleinement attaché à ce que les outils qui servent chaque jour les acheteurs publics soient adaptés à leurs besoins et à leurs pratiques. À cette

et nombreux. Le projet de PNAAPD est mis en consultation publique. Au moment où je vous parle, il est disponible en ligne. Je vous invite à répondre à cette consultation en tant que parlementaires

robuste. Cette évolution, loin d'être superficielle, ne peut être ajoutée sans concertation préalable avec l'ensemble des parties prenantes et, surtout, sans étude d'impact juridique poussée.

la portée des trois grands principes constitutionnels de la commande publique, énoncés à l'article L. 3 du code de la commande publique. Toutefois, la référence aux ODD dans la commande publique figure désormais dans un article L.

en l'état le droit actuel concernant la prise en compte des objectifs de développement durable. Actuellement, dans le cadre d'un marché, l'acheteur doit prendre en compte les ODD dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. L'article 15 prévoit d'ajouter une obligation écrite venant justifier l'accomplissement de cette obligation. Cette disposition ne semble pas pertinente. En effet, elle vient ajouter une obligation supplémentaire ne permettant pas d'atteindre les ODD en tant que tels. L'ajout de nouvelles règles risque de nuire à l'efficacité économique et à la mise en oeuvre de l'action publique. Ainsi, cet amendement tend à supprimer l'obligation de justification relative à la prise en compte des ODD afin

: La parole est à M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à assurer la prise en compte d'objectifs environnementaux dans les marchés relevant de la commande publique, dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des travaux, fournitures ou services objets du marché. Les marchés publics représentent environ 8 % du PIB de la France. Pour autant, selon l'Observatoire économique de la commande publique (OECP), seuls 10 % des contrats comportaient des clauses environnementales en 2018. Cet amendement vise à fixer comme objectif de limiter l'impact environnemental des commandes L'article L. 2124-2 du code de la commande publique régit la procédure d'appel d'offres et appelle l'acheteur public à faire le choix de l'« offre économiquement la plus avantageuse La Convention citoyenne pour le climat a souligné la nécessité de renforcer les clauses environnementales dans le passage de marchés publics, pour répondre aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre et pour engager une véritable transition énergétique et écologique dans les secteurs qui relèvent de l'action publique. Cet amendement vise à allier enjeux écologiques et économiques en donnant aux acheteurs publics la possibilité de choisir l'offre la plus avantageuse économiquement parmi les offres ambitieuses écologiquement, sans que cela soit en contradiction avec les critères économiques. Enfin, il tend à limiter à un an le délai d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux marchés publics. En effet, si le délai doit permettre l'adaptation aux nouvelles mesures, les marchés en cours ne sont pas concernés

Les marchés publics constituent à la fois un levier financier fort pour réaliser la transition et un symbole pour encourager la transformation de la société. Introduire systématiquement des clauses environnementales dans les marchés publics permettra de favoriser les entreprises vertueuses et des achats plus locaux et durables. Par ailleurs, cela incitera d'autres entreprises à s'engager également dans ce sens. Aussi les modifications proposées par l'article 15 sont-elles les bienvenues. Cet amendement vise à introduire la durabilité comme critère de discrimination des offres dans le cadre des marchés publics, aux côtés des critères économiques.

En ajoutant le critère social comme alternative au critère environnemental, l'amendement adopté en commission affaiblit l'ambition initiale du Gouvernement en matière environnementale.

la plus avantageuse économiquement. Vous avez pour votre part choisi de retenir la formulation générale de « caractéristiques environnementales ou sociales » pour préserver la liberté des acheteurs de choisir les critères à retenir. Or une telle approche est moins ambitieuse et ne constitue pas un signal suffisamment fort sur l'importance de la transition écologique dans la commande publique. Ce manque d'ambition bouche l'horizon d'une commande publique immédiatement environnementale. Il n'est pas urgent d'attendre, il est urgent d'agir. d'agir. On nous oppose que le droit européen ne permet pas de promouvoir l'offre écologiquement la plus avantageuse au même niveau que l'offre économiquement la plus avantageuse. Pour notre part, nous pensons que notre pays doit être le fer de lance de cette évolution de la commande publique.

pour les marchés de travaux, de services et de fournitures. Cette évolution permettra de concrétiser les objectifs des pouvoirs publics en faveur de la transition écologique. Le délai maximal de cinq ans prévu au II de l'article 15

Il serait ainsi pertinent de prévoir une mise en oeuvre plus rapide des obligations pour les concessions et délégations, dont les durées d'exécution sont généralement plus longues que celles des marchés publics. En revanche, pour certains marchés de prestations intellectuelles, l'inclusion de considérations environnementales pourra demander un travail de réflexion plus approfondi.

prévoit que la commande publique doit prendre en considération des données environnementales pour l'attribution des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Cette orientation va dans le bon sens et je la partage.

Comme l'a rappelé le Conseil d'État dans son avis, le concept d'« offre la plus avantageuse écologiquement et économiquement » serait contraire au droit de l'Union européenne. L'autre solution trouvée dans le projet de loi- imposer la prise en compte d'un critère environnemental dans l'attribution du marché -répond à cette préoccupation, sans poser de difficultés au regard du droit européen. Par ailleurs, il semble irréaliste de prévoir une entrée en vigueur des dispositions de l'article 15 relatives aux marchés publics

Les dispositions sur lesquelles le Gouvernement souhaite revenir par cet amendement ne posent pas de difficultés au regard du droit de l'Union européenne et permettent de concilier considérations environnementales et sociales. n° 802, pour des raisons que j'ai précédemment invoquées. Le concept d'« offre la plus avantageuse écologiquement et économiquement » ne peut pas être retenu en raison du droit européen.

d'entrée en vigueur des dispositions relatives au verdissement des marchés publics, compte tenu notamment de l'hétérogénéité de ces marchés. En tout état de cause, l'entrée en vigueur pourra être anticipée par voie réglementaire, comme l'a rappelé le Conseil d'État. Quel est l'avis du Gouvernement

même argument que le rapporteur. J'ajoute que la prise en compte du cycle de vie des travaux, des fournitures et des services objets du marché est déjà spécifiquement prévue en droit à l'article L. 2112-3 du code de la commande publique parmi les clauses d'exécution. C'est pourquoi le

de voir les TPE-PME et les artisans accéder plus facilement aux marchés publics ; ceux-ci peuvent d'ailleurs déjà bénéficier d'outils favorisant leur accès aux contrats publics grâce à l'allotissement, à l'autorisation des variantes ou encore aux conditions favorables de versement d'avances financières. Il n'est cependant pas juridiquement possible de prévoir dans la loi que les marchés doivent être attribués selon des critères différents en fonction de la taille des entreprises. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement

de l'offre économiquement la plus avantageuse ni à la condition que les critères d'attribution soient objectifs, précis, liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, le respect de ces règles étant imposé

des achats publics socialement et écologiquement responsables, les Spaser, dans le but d'inscrire la politique d'achat dans une démarche de durabilité des produits, d'efficacité énergétique et de sobriété. Ces moyens d'action ont été identifiés dans la stratégie nationale bas-carbone. L'achat public doit jouer un rôle clé et vertueux dans la relance.

et à mieux intégrer l'enjeu de durabilité des produits et de sobriété dans leurs actions.

deux siècles une gouvernance démocratique entre sociétaires, qui ne nie pas les spécificités professionnelles ou hiérarchiques et qui reconnaît à chaque travailleur ou sociétaire une capacité d'intervention dans la gestion de l'entreprise. Il s'agit donc d'inclure ces modes de gouvernance à la fois innovants et et démocratiques dans les secteurs promus par les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. L'amendement

que celle de profits financiers, justifie de renforcer la place des entreprises sociales et écologiques dans les Spaser. Les avantages de ces modes de gouvernance, en particulier dans le secteur énergétique, sont d'ailleurs reconnus par la Commission européenne, qui a récemment introduit dans le droit européen les « communautés énergétiques », régies par des modes de gouvernance démocratique. Il convient donc de renforcer le rôle des Spaser en favorisant l'ancrage et les retombées sur le territoire, l'intégration des parties prenantes et les modes de gouvernance innovants. Les

sur tout le territoire français : laveuses, équipements pour le transport et la logistique, parcs d'emballage et de caisse, adaptation des lignes de conditionnement, communication et affichage dans les lieux de vente. Si ces infrastructures sont créatrices d'emplois et, à terme, moins coûteuses que la gestion des déchets d'emballages jetables, elles requièrent néanmoins un investissement initial qui peut être important pour certains acteurs. à l'économie circulaire (AGEC) prévoit qu'au moins 2 % des écocontributions perçues par l'éco-organisme chargé des emballages doivent être consacrés au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages. Ces financements pourraient être complétés par une commande publique exemplaire privilégiant les dispositifs de réemploi des emballages et orientant ainsi les investissements des acteurs. Cet amendement vise donc à orienter les acheteurs publics vers des dispositifs de réemploi des emballages, lorsque cela est possible. Cet amendement a été travaillé avec l'ONG Zero Waste France et le Réseau Action Climat.

Il nous semble indispensable de réorienter les acheteurs publics vers des dispositifs de réemploi des emballages, qui permettent d'économiser des matériaux et de créer des filières. La loi AGEC prévoit déjà d'ailleurs l'obligation pour l'État d'acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Le décret d'application de cette mesure a été pris le 9 mars dernier. Il comporte en annexe un tableau dans lequel figure l'intégralité des produits issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, pour lesquels sont fixées des proportions minimales annuelles d'achat. Toutefois, ce décret, en son tableau annexe, prévoit une part encore trop peu importante de réemploi. Ainsi, celle-ci s'élève à seulement 20 % pour les sacs d'emballage, dont 10 % sont strictement issus du réemploi et de la réutilisation,

Pourtant, comme le souligne le Réseau Action Climat, que nous avons auditionné, le réemploi des emballages présente un bilan écologique favorable. En amont, il évite l'extraction de nouvelles ressources, sachant que les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et de plus de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique. En aval, il permet de diminuer le nombre d'emballages à recycler, à incinérer ou à enfouir. Ce sont autant de pollutions liées à ces modes de traitement qui sont évitées. De plus, les filières de réemploi participent à la redynamisation des économies locales par la création d'emplois non délocalisables, notamment une partie en insertion.

sur la généralisation de la consigne pour les emballages en verre, cet amendement vise à orienter la commande publique vers des dispositifs de réemploi des emballages. Les services de l'État et les collectivités territoriales devront privilégier, avec une échéance raisonnable fixée à 2025, les solutions de réemploi des emballages, lorsque cela est possible, pour leurs achats publics.

ne sont qu'au début de leur évolution. La commande publique pourrait compléter les 2 % d'écocontribution fixés dans la loi AGEC pour le développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages. Ainsi, mes chers collègues, le développement de la filière de réemploi des emballages, en tant qu'alternative vertueuse aux emballages jetables, nécessite des investissements et des financements à la hauteur, notamment pour construire les infrastructures nécessaires. La commande publique a ici pleinement son rôle à jouer. Quel est l'avis de la commission ? La

sur les amendements n 1475 et 406. Il ne semble pas non plus nécessaire de préciser que les Spaser concourent au développement des modes de gouvernance de l'économie sociale et solidaire.

outre, rien ne justifie de compléter l'article relatif aux Spaser d'un objectif spécifique sur les emballages réemployables, alors qu'il ne prévoit par ailleurs aucun objectif précis. Enfin, la commission émet un à préciser que les solutions de réemploi des emballages doivent être privilégiées par l'État et les collectivités territoriales. Ces amendements sont de fait satisfaits par la loi AGEC, qui prévoit des dispositions relatives au réemploi dans la commande publique.

pour rédiger leurs cahiers des charges. Cette clause, qui prévoit non seulement le réemploi des emballages, mais aussi le caractère recyclable des matériaux d'emballage, est applicable et effective depuis le 1 avril dernier. Comme l'a indiqué le rapporteur, les dispositions du décret du 9 mars dernier pris en application de la loi AGEC prévoient d'ores et déjà l'obligation pour les acheteurs publics d'acquérir une proportion de produits issus du réemploi ou de la réutilisation. Ces amendements étant satisfaits, le Gouvernement en demande leur retrait ; à défaut, il

Afin de faire des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, les Spaser, de véritables leviers en faveur d'une commande publique locale plus durable, il paraît opportun d'intégrer des indicateurs précis concernant les catégories d'achat socialement et écologiquement responsables. La mise en oeuvre d'une publication régulière de ces indicateurs est également souhaitable pour que les bonnes pratiques puissent essaimer. En outre, la publication et le suivi d'indicateurs sont indispensables pour permettre d'évaluer les politiques de l'achat public.

Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur [ ...] adopte un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » Ce schéma contribue également à la promotion d'une économie circulaire.

l'avis de la commission ? Si l'introduction d'indicateurs précis concernant les catégories d'achats socialement et écologiquement responsables dans les Spaser semble opportune pour faire de ces derniers de véritables leviers en faveur d'une commande publique locale plus durable, une publication annuelle

les avancées introduites en première lecture à l'Assemblée nationale sur les Spaser en les complétant d'une obligation d'inclusion d'un objectif spécifique sur les dépenses ou marchés confiés à des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail et par des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables. Quel est

Lahellec. L'article 15 prévoit que les contrats liés à la commande publique prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. Pour autant, nous estimons que l'introduction d'un critère évaluant l'impact carbone dans le transport d'un produit en renforcerait la spécification de la qualité écologique. Cela renvoie

la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre fait déjà pleinement partie des objectifs de l'article 15. Toutefois, cet article ne saurait comprendre une énumération de l'ensemble des considérations environnementales susceptibles d'être prises en compte dans les conditions d'exécution en fonction de l'objet du marché.

lors de la passation de marchés de travaux, de services ou de fournitures. Acheter local en fait à l'évidence partie. Cet amendement, qui a échappé à la guillotine de l'article 45 de la Constitution, vise à ajouter un caractère local aux critères que devra prendre en compte de manière obligatoire la commande publique dans la rédaction et la sélection des appels d'offres. Vous l'avez compris, il s'agit de favoriser les circuits courts et le caractère local des productions, afin d'encourager les entreprises de proximité, par définition moins émettrices de carbone.

transition écologique nécessitent des approches transversales et des coopérations innovantes entre acteurs privés et publics sur les territoires. Ces acteurs, tout particulièrement ceux de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire, proposent des consortiums et des solutions intégrées dont les avantages sont actuellement insuffisamment perçus ou valorisables par la commande publique. Actuellement, les « coûts évités » ne sont en effet pas, ou très peu, pris en compte par les collectivités locales lors de l'examen des mémoires techniques et des propositions financières en réponse aux appels d'offres et appels à projets, alors que les candidats proposent des solutions et coopérations permettant de réduire les coûts financiers et écologiques dans la mise en oeuvre des moyens et prestations objets de la commande. vise à faire en sorte que la commande publique prenne en compte la notion de coûts évités mis en avant par ces coopérations et l'intègre systématiquement parmi les critères de notation des réponses aux appels d'offres et appels à projets. à projets. Il s'agit d'ajouter les coûts évités en matière financière et écologique à la liste des considérations prises en compte dans les commandes publiques, en particulier dans la notation de la qualité des mémoires techniques. Un recours plus important à la procédure des « variantes » dans les cahiers des charges de la commande publique pourrait également soutenir le développement des coopérations et innovations territoriales et la prise en compte des coûts évités.

Demilly. Cet amendement a pour objet d'inclure l'économie circulaire parmi les considérations prises en compte pour apprécier les conditions d'exécution des marchés publics. Dans l'optique d'un verdissement de la commande publique, l'économie circulaire réduit à l'évidence l'usage des matériaux et la consommation d'eau et d'énergie. Son incorporation au principe d'exécution des marchés contribuerait donc à la mise en oeuvre de stratégies respectueuses du climat.

contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation. Aujourd'hui, les apprentis et les personnes en contrat de professionnalisation ne sont pas systématiquement pris en compte dans la liste des personnes éligibles aux actions d'insertion. Or le contrat d'apprentissage et le contrat de objet même dans le code du travail, contribuent tous deux à l'insertion professionnelle. Leur prise en compte est d'autant plus importante dans le contexte actuel de crise sanitaire. Elle s'inscrit dans le plan de relance « 1 jeune, 1 solution », lancé

que le taux d'insertion dans l'emploi des contrats d'alternance est très fort. Cela répond pleinement à l'objectif d'insertion fixé par le législateur. Quel est l'avis de la de la commission ? Cet amendement vise à faire en sorte que les bénéficiaires de contrats d'alternance soient pris en compte lorsque les conditions d'exécution prévoient des considérations relatives à l'insertion sociale. Un tel ajout me semble imprécis et source de confusion. Il est susceptible de créer des incertitudes pour les acheteurs publics, notamment pour nos collectivités territoriales. La commission émet donc un avis défavorable

défavorisées de retrouver des conditions de leur intégration dans le monde professionnel. Si les contrats d'alternance constituent un outil efficace de l'intégration des jeunes en entreprise, ils ne s'adressent pas spécifiquement à des personnes en difficulté. Pour ces raisons, comme pour celles qui ont été mises en avant par M.

ainsi de faire de la commande publique un levier d'inclusion et de cohésion sociale. Il est également proposé que les marchés de travaux et services passés selon une procédure formalisée prévoient une part minimale que le titulaire s'engage à confier aux soumissionnaires affectant des personnes vulnérables à l'exécution du marché, en particulier à travers des structures d'insertion par l'activité économique. Toute impossibilité à mettre en oeuvre cette obligation devra être justifiée. Cet amendement, en lien direct avec les objectifs de justice sociale et de verdissement de l'économie du projet de loi, est issu d'un travail avec la fédération des entreprises d'insertion et Alliance Villes Emploi.

des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables me semble contraire au droit de l'Union européenne. Je suis très sensible aux problématiques d'inclusion, mais je ne peux pas prendre le risque de voir l'ensemble des marchés publics passés par nos collectivités territoriales

du Gouvernement ? Si les marchés de travaux et de services d'un certain montant peuvent être des vecteurs privilégiés pour favoriser l'insertion professionnelle des publics en difficulté, il ne paraît pas pertinent d'en faire une obligation légale. Tous les marchés visés ne s'y prêtent pas nécessairement, notamment lorsque la durée d'exécution du contrat n'est pas suffisante pour mettre véritablement en place les parcours d'insertion professionnelle ou lorsqu'il est impossible de justifier d'un lien

en fonction des spécificités de leurs achats, les caractéristiques des secteurs d'activité et les modalités de mise en oeuvre des objectifs en matière sociale dans la commande publique. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

: La parole est à M. Hervé Gillé. Le texte adopté à l'Assemblée nationale comportait un dispositif visant à favoriser le développement des entreprises solidaires d'utilité sociale. première, les alinéas 11 à 15 de l'article 15 prévoyaient ainsi que les marchés ayant un objectif écologiquement responsable devaient prévoir la part minimale de l'exécution du marché que le titulaire s'engageait à confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées ou à des structures équivalentes. Cette part ne pouvait pas être inférieure à 5 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permettait pas. Les travaux de la commission ont abouti à la suppression d'un tel dispositif. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain considère au contraire une telle mesure comme une avancée significative. Nous sommes en effet encore loin des objectifs fixés dans le cadre du pacte d'ambition pour l'insertion par l'activité économique, à savoir stimuler les clauses sociales,

Nous proposons donc non seulement de rétablir le dispositif dans le texte, mais également d'ajuster la part minimale d'exécution d'un marché à confier à une entreprise solidaire à 10 % du montant prévisionnel du marché, au lieu des 5 % prévus par les députés. souhaitons qu'un décret fixe un seuil d'application pour déterminer les marchés concernés par une telle mesure.

(ESUS) ou à des structures équivalentes est manifestement contraire au droit de l'Union européenne. Nous avons eu l'occasion de le rappeler en commission avec le rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission émet donc un avis défavorable

de retirer ces alinéas pour sécuriser les marchés.

il paraît prématuré de modifier le cadre législatif relatif au devoir de vigilance. Le Parlement européen a d'ailleurs fait usage de son droit d'initiative législative et adopté une position officielle le 10 mars 2021- c'est donc d'actualité -sur le devoir de vigilance, enjoignant ainsi à la Commission européenne de produire un projet de législation. Dans ce contexte, il paraît donc inutile de surjouer les bons élèves, au risque de créer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises françaises. L'amendement

pour l'acheteur public d'écarter d'un marché public les grandes entreprises qui n'ont pas publié de plan de vigilance. Il s'agit simplement d'inciter les acteurs économiques à appliquer la loi. C'est

Si les entreprises françaises se saisissent suffisamment tôt de cette obligation, elles disposeront sans aucun doute d'un avantage par rapport à leurs concurrentes européennes, qui seront moins préparées à l'application de ce nouveau cadre juridique. Telles étaient d'ailleurs les conclusions d'un récent rapport du Conseil général de l'économie.

pour l'acheteur public d'écarter d'un marché public les grandes entreprises qui n'ont pas publié de plan de vigilance. Il s'agit simplement d'inciter les acteurs économiques à appliquer la loi. C'est donc bien un cadre facultatif, et non obligatoire.

Le verdissement de l'économie souhaité par le projet de loi s'accompagne de la volonté du renforcement de la justice sociale, pour faire rimer économie verte avec économie inclusive. C'est pourquoi il serait vertueux de valoriser les soumissionnaires qui affectent à la réalisation des marchés des personnes défavorisées, afin d'encourager la diffusion de pratiques inclusives dans toute l'économie. amendement est directement inspiré par le considérant 99 de la directive européenne du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, selon les mesures visant à [ ...] favoriser l'intégration des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables parmi les personnes chargées d'exécuter le marché, ou à former aux compétences nécessaires pour le marché en question, peuvent également faire l'objet de critères d'attribution ou de conditions d'exécution du marché, à condition d'être liées aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché Les modalités de la bonification resteront à déterminer par voie réglementaire. Il s'agit non pas de mettre en place des quotas ou de refuser des marchés à toute entreprise n'incluant pas ce facteur social,

reviendrait à poser une obligation de prise en compte d'un critère social dans l'attribution de l'offre. Or il est très difficile d'envisager que tous les marchés publics soient liés à des critères sociaux.

est ainsi libellé : La parole est à M. Henri Cabanel. Cet amendement vise à intégrer les structures de l'insertion par l'activité économique à l'article L. 2152-9 du code de la commande publique, qui renforce l'accès des PME et des artisans aux marchés globaux en obligeant les acheteurs publics à prévoir un critère tenant compte des engagements des candidats à leur réserver une part de l'exécution de ces marchés. Il s'agit ainsi de valoriser les candidatures des soumissionnaires qui prévoient de sous-traiter une partie de l'exécution du marché à ces structures, afin de permettre aux salariés en insertion de bénéficier de passerelles vers un emploi durable. Quel est l'avis de la commission ?

contribue également à soutenir les publics vulnérables, pour qui le passage au sein de l'entreprise constitue une étape indispensable du parcours d'insertion. Ces entreprises concourent donc à la réalisation des objectifs du projet de loi, dans ses aspects tant environnementaux que sociaux.

La nouvelle disposition englobe ainsi les entreprises inclusives dans la part PME existante. Comme l'a fort justement rappelé le rapporteur lors de l'examen en commission, la « dérogation aux règles de la commande publique pour par l'objectif d'intérêt général visant à corriger une inégalité entre ces entreprises aux moyens limités et les plus grandes entreprises, permettant ainsi de rejoindre l'objectif d'égal accès à la commande publique et de concurrence C'est davantage le cas encore des entreprises qui intègrent de façon importante des personnes en difficulté, comme les entreprises adaptées. Lorsqu'elle est majoritaire dans les effectifs de l'entreprise, cette intégration représente en effet un surcoût par rapport à l'intégration de collaborateurs non défavorisés- moindre productivité, surencadrement technique nécessaire, dimension sociale à intégrer dans le service des

de l'amendement n° 1490 ferait, elle aussi, courir un risque juridique aux acheteurs dès lors que cela permettrait, en méconnaissance du droit européen et des principes constitutionnels, de privilégier des entreprises en fonction de leur finalité, leur mode de fonctionnement ou leur politique générale. En outre, les entreprises de l'économie sociale et solidaire bénéficient déjà de l'article L. 2113-15 du code de la commande publique, expressément autorisé par le droit européen, qui permet aux acheteurs de leur réserver l'attribution de certains

Ces acteurs, tout particulièrement ceux de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire, proposent des consortiums et des solutions intégrées dont les avantages sont insuffisamment perçus ou valorisables actuellement par la commande publique. publique. Cette économie devrait pouvoir faire l'objet d'une préférence des collectivités, de plus en plus soucieuses de leur responsabilité environnementale, y compris dans leurs commandes publiques. Actuellement, les coûts évités ne sont pas ou peu pris en compte par les collectivités locales lors de l'examen des mémoires techniques et des propositions financières en réponse aux appels d'offres et appels à projets, alors que les candidats, souvent acteurs de l'économie sociale et solidaire, proposent des solutions et coopérations permettant de réduire les coûts financiers et écologiques dans la mise en oeuvre des moyens et prestations objets de la commande. L'objectif de cet amendement est que la commande publique prenne en compte la notion de coûts évités mis en avant par ces coopérations et l'intègre systématiquement parmi les critères de notation des réponses aux appels d'offres et appels à projets. Son inscription dans la loi permettra de reconnaître les avantages à long terme d'une commande publique soucieuse de son impact et de son coût sur l'environnement. Aucune obligation n'incombera pour autant aux collectivités, qui resteront libres dans leur choix, mais auront à leur disposition beaucoup plus de latitude pour

comme alternative aux clauses et critères environnementaux, l'amendement adopté en commission remet en cause l'obligation initiale de prendre en compte de façon obligatoire les considérations environnementales

M. Daniel Salmon. Sur l'initiative du Sénat, la loi AGEC a fixé un objectif national de réemploi équivalent à 5 % du poids des déchets ménagers à l'horizon 2030. De ce fait, la France a été le quatrième pays européen à s'appliquer un objectif national de réemploi, après l'Espagne, la Belgique et la Suède ; nous pouvons nous en féliciter. Cet objectif s'applique à l'État et aux collectivités territoriales et doit être décliné au sein des filières à responsabilité élargies des producteurs, mais seul ce dernier aspect est précisé dans la loi. Cela se révèle dommageable. En effet, aucune communication du Gouvernement ou des services de l'État ou des collectivités territoriales n'a rappelé ou promu cet objectif. Le ministère de la transition écologique omet même de le citer dans ces fiches traitant du réemploi.

Cet amendement vise donc à clarifier utilement l'intention du Sénat exprimée en 2019. À l'heure de l'épuisement de nos ressources primaires et stratégiques, le développement du réemploi est un enjeu majeur pour nos sociétés. Il est indispensable que l'ensemble des pouvoirs publics, qu'ils soient centraux ou déconcentrés, y participent activement

Dans les échanges avec les parties prenantes qui ont précédé l'élaboration de ce projet de loi, le délai de mise en oeuvre de cinq ans pour tous les marchés a recueilli un consensus. Cet amendement tend à le maintenir. La parole est à M.

afin de donner aux autorités concédantes et aux entreprises le temps minimum nécessaire pour adapter leurs méthodes d'achat et leurs offres. Réduire ce délai maximal à deux ans paraît difficilement atteignable et emporterait des inconvénients allant à l'encontre de l'objectif.

à la rédaction du texte adoptée par l'Assemblée nationale. Cette partie de l'article 15 doit pouvoir entrer en vigueur dans les meilleurs délais, mais cette application doit se faire avec méthode, rigueur et dialogue. Ainsi, pour les contrats de concession comme pour les marchés publics, il est nécessaire d'engager une consultation de l'ensemble des acteurs pour identifier leurs contraintes et leurs besoins. Seule cette consultation permettra de déterminer le temps nécessaire aux entreprises et aux acheteurs pour s'adapter à de nouvelles normes qui peuvent nécessiter une réorganisation importante de leurs méthodes de travail, notamment pour les PME ou les associations titulaires de délégation de services publics locaux, en particulier dans les secteurs du tourisme, des installations sportives, de l'accueil périscolaire, des services culturels ou du transport de voyageurs. C'est pourquoi ce délai de cinq ans nous paraît nécessaire.

considéré que les soumissionnaires à des contrats de concession sont généralement- je prends soin de le dire avec toutes les précautions d'usage -des entreprises d'une taille plus importante que celles qui répondent à des marchés publics. Un délai d'entrée en vigueur ramené à deux ans en matière de contrats de concession

Pour les contrats de concession comme pour les marchés publics, il est nécessaire d'engager une consultation de l'ensemble des acteurs pour identifier les contraintes et les besoins. Elle seule permettra de déterminer avec précision le temps nécessaire aux entreprises comme aux acheteurs pour s'adapter à des contraintes nouvelles qui peuvent nécessiter une réorganisation de leurs méthodes de travail, notamment pour les PME ou les associations titulaires de délégation de services publics locaux, en particulier dans les secteurs du tourisme, des installations sportives, de l'accueil périscolaire, des services culturels ou encore du transport de voyageurs. Un délai d'entrée en vigueur de ces mesures inférieur à cinq ans pour les contrats de concession présenterait un risque important que les obligations soient mises en oeuvre de manière incomplète ou bancale et que les entreprises se détournent de la commande publique. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur ces trois amendements. Je mets aux voix

C'est une lapalissade de dire que le recours aux circuits courts permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or le droit de la commande publique ne permet pas suffisamment aux élus locaux, spécifiquement aux maires, de soutenir les entreprises de proximité. Cet amendement vise donc, de façon audacieuse- j'en conviens -, à dispenser de mise en concurrence l'acheteur qui se fixe un objectif écologiquement responsable dans le respect des seuils réglementaires de droit européen sur la passation des marchés publics. C'est audacieux, en effet ! L'article L. 2122-1 du code de la commande publique définit les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à l'obligation de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables. La méconnaissance de ce principe fondamental de la commande publique doit être strictement proportionnée. Il me semble que la poursuite d'un « objectif écologiquement responsable » ne constitue pas un motif suffisant, notamment au regard du caractère particulièrement vague de cette expression. l'avis du Gouvernement

visant un « objectif écologiquement responsable » porte atteinte aux principes de la commande publique- liberté d'accès, égalité de traitement et transparence -qui s'imposent, sous réserve de quelques dérogations extrêmement limitées, dès le premier euro.

Concrètement, cela signifierait par exemple qu'une collectivité territoriale pourrait, pour un marché de fournitures, se dispenser de formalisme jusqu'à 214 000 euros, dès lors qu'elle viserait un objectif écologiquement responsable. Il s'agit là encore de soutenir nos entreprises de proximité et de favoriser une consommation locale et respectueuse de l'environnement. est l'avis de la commission ? Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché dans le respect des principes de la commande publique. Il est possible de passer un marché selon une procédure adaptée, notamment lorsque la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure à des seuils fixés par le droit européen- vous l'avez rappelé. cet amendement me semble poser deux difficultés principales. D'une part, la possibilité de passer un marché selon une procédure adaptée serait ouverte dès lors que le marché vise « un objectif écologiquement responsable ». Or cette formulation est assez vague. autre écueil, il est précisé que l'acheteur pourrait alors adapter librement les modalités de publicité du marché. Or cette formulation pourrait être attentatoire aux principes fondamentaux de la commande publique. En conséquence, la commission sollicite l'avis du Gouvernement.

dont la valeur estimée est supérieure à 90 000 euros. Cette publicité obligatoire contribue directement à la transparence des procédures, mais aussi à un meilleur accès des entreprises à la commande publique, en centralisant les avis de publicité. Il s'agit non d'un formalisme inutile,

: La parole est à M. Joël Guerriau. Présenté comme un outil au service de la transition énergétique, le numérique est de plus en plus mobilisé dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques publiques, notamment en matière d'aménagement du territoire et de transport public. Toutefois, toutes les solutions numériques ne génèrent pas un gain environnemental. Construire un système numérique résilient implique de choisir des solutions dont l'impact carbone est positif. Il est donc proposé que l'impact environnemental des solutions numériques pour toute leur durée de vie soit systématiquement pris en compte dans l'évaluation des offres présentées par les candidats à un marché public.

Bigot. Présenté comme un outil au service de la transition énergétique, le numérique est de plus en plus mobilisé dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques publiques. Toutefois, les solutions numériques ne génèrent pas forcément un gain environnemental. Notre objectif est de garantir la convergence entre transition écologique et transformation numérique et de veiller à ce que la seconde soit bien un accélérateur de la première. Nous sommes encore peu outillés pour faire de l'environnement un facteur déterminant dans nos choix politiques. La France manque d'outils et d'indicateurs partagés pour mesurer les impacts environnementaux du numérique et ainsi mieux cibler les actions à mettre en oeuvre prioritairement. Nous avons besoin de progresser collectivement sur l'évaluation environnementale de ce que nous mettons ou mettrons en place. Aussi, lorsqu'ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs doivent tenir compte des incidences environnementales de cette solution.

l'avis du Gouvernement ? C'est un peu le même débat que celui que nous avons eu précédemment sur le carbone dans les transports. Faut-il ou non spécifier l'intégralité des volets

de prendre en compte les considérations liées aux aspects environnementaux des travaux, des services et des fournitures qui sont achetées. Certes, ces amendements

européen. Les panneaux photovoltaïques chinois sont certes vendus à des prix relativement bas, mais leur production a, en plus d'être le fruit de conditions de travail discutables et de salaires particulièrement bas, des conséquences environnementales importantes. On constate en effet des rejets massifs dans l'atmosphère de poudre de silicium et une pollution désastreuse

Par ailleurs, ces panneaux ont un bilan carbone peu intéressant, une durée de vie qui n'est pas optimale et des capacités de valorisation et de recyclage relativement faibles. Au vu de ces enjeux environnementaux et sanitaires, il semble important de prendre en compte le bilan carbone et environnemental sur l'ensemble de la chaîne de production des panneaux photovoltaïques achetés par la commande publique. Par ailleurs, il existe en France une production de silicium, des fabricants de modules photovoltaïques et des entreprises qui produisent intégralement des panneaux solaires, parfois totalement recyclables. Victimes du dumping social et environnemental et de la concurrence chinoise, ces entreprises sont souvent en difficulté la France dispose de tous les atouts pour développer une filière solaire puissante, lui permettant d'accroître sa souveraineté et sa résilience, comme le propose l'intitulé de ce projet de loi. Pour permettre son développement, la puissance publique doit l'accompagner. Favorisé dans la commande publique, l'achat de panneaux photovoltaïques photovoltaïques aux caractéristiques environnementales exigeantes est une manière de se tourner vers les productions françaises et européennes. Cela s'inscrit dans la philosophie de ce projet de loi, comme dans celle de la loi AGEC qui a voulu favoriser l'emploi de matériaux biosourcés dans la commande publique. Quel est l'avis de la commission

le réemploi et le recyclage des panneaux photovoltaïques, ainsi que leur impact environnemental en analyse de cycle de vie. C'est un sujet particulièrement important et il me semble pertinent que la commande publique puisse s'en saisir. Je note toutefois que la formulation de l'amendement est quelque peu vague

place avec l'aide de l'Ademe. Je suppose que ce type de dispositif perdure. De ce fait, une entreprise qui présentait un dossier avec des panneaux photovoltaïques fabriqués en Chine avait nécessairement un bilan carbone bien plus mauvais

n° 3 rectifié . La commande publique désigne les contrats passés par les collectivités territoriales, l'État et les établissements publics, ainsi que leurs groupements. Représentant plus de 8 % du PIB, elle est un levier majeur de mise en oeuvre des politiques publiques. regard à la fois de la nécessité de relance d'une économie favorable à une économie circulaire, du rôle d'exemplarité de l'État et des nombreuses obligations imposées aux acheteurs publics, issues notamment de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, il importe d'aider ces acteurs de manière opérationnelle à intégrer des aspects de cette nouvelle économie dans leurs achats. dans leurs achats. L'État devra mettre à disposition des acheteurs publics des outils de définition du coût du cycle de vie pour les différents segments d'achat- fournitures, parc automobile, immobilier, informatique et télécommunications afin d'accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la définition de leur politique d'achat et de les éclairer dans leur prise de décision. Ces outils devront intégrer le coût global lié à l'acquisition, à l'utilisation, à la maintenance et à la fin de vie, ainsi que les coûts externes supportés par l'ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, l'émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. Cet objectif pour 2022 a été inscrit dans la feuille de route pour une économie circulaire. Il s'agit aujourd'hui de s'assurer de sa réalisation.

Il s'agit de faire en sorte que l'État mette à disposition des acheteurs publics des outils de définition du coût du cycle de vie pour les différents segments d'achat, afin d'accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la définition de leur politique d'achat et de les éclairer dans leur prise de décision. Nombre d'adjudicateurs locaux se sont déjà emparés des possibilités d'inclure des critères plus respectueux de l'environnement et de la biodiversité. Pour autant, leur capacité à évaluer ce qui relève d'une démarche vertueuse ou non peut être limitée et cette évaluation peut se révéler différente d'une collectivité à une autre. Aussi, dans un souci de cohérence et pour pallier les insuffisances d'ingénieries locales disparates, nous souhaitons, par cet amendement, que l'État mette à disposition des outils pratiques pour définir les coûts, que ce soit en matière d'émission de CO2, de perte de biodiversité ou de déforestation, du cycle de vie des différents achats. Comme toujours, une meilleure information permet de meilleures décisions. La commande publique entrant pour près de 8 % dans notre PIB, ce levier majeur de verdissement de l'économie doit être au coeur de notre attention. Quel

Outil essentiel de la mesure de l'efficacité de la valorisation des activités et des politiques publiques, la comptabilité doit prendre en compte les enjeux écologiques pour transformer sur le fond les indicateurs de performance de notre pays. Il est donc proposé que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les possibilités de mise en place, à terme, d'une comptabilité publique et privée écologique.

2022 est prévue l'obligation pour les acheteurs publics d'acquérir des biens issus du réemploi : 20 % de leurs téléphones, 30 % de leurs pneumatiques rechapés,

commission ? En application de la loi AGEC, le décret du 9 mars 2021 est venu fixer des obligations d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation dans un certain nombre de cas.

Nous cherchons à compléter la transposition du règlement du Parlement européen du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Ce règlement prévoit de nouvelles obligations à la charge de certaines entreprises du secteur, dont le respect doit être contrôlé par les autorités nationales compétentes, conformément à la législation sectorielle applicable. Pour ce qui concerne les sociétés de gestion, le code monétaire et financier dispose que l'Autorité des marchés financiers (AMF) veille à la qualité de l'information fournie. revanche, pour toutes les autres entités visées, notamment les entreprises d'assurance et de réassurance, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la Caisse des dépôts et consignations, les mutuelles et unions, les institutions de prévoyance et leurs unions, ainsi que les institutions de retraite professionnelle, rien n'est prévu

L'évolution concomitante du droit européen, dont nous avons parlé, et du droit national en matière de finance durable aura des conséquences importantes sur le périmètre et le champ de contrôle de l'ACPR sur ses assujettis. J'ajoute les exigences en matière de extrafinancier qu'emportent le règlement européen et le décret récemment publié, qui vient revisiter le dispositif issu du VI de l'article croissance verte. Le Gouvernement accueille positivement l'extension des pouvoirs du superviseur bancaire et assurantiel en la matière. C'est une évolution bienvenue-